relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de mener une mission d'information sur les dysfonctionnements constatés dans l'organisation des élections départementales et régionales de juin 2021.

de la commission des lois. En conséquence, la commission des lois se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information. Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié.

qui, dois-je le rappeler, fixe des limites aux possibilités offertes par les progrès de la recherche. Concilier le possible et le souhaitable, voilà la mission délicate qui est la nôtre, la vôtre comme celle du Gouvernement, dans les débats qui nous réunissent depuis bientôt deux ans sur ce texte. L'assistance médicale à la procréation (AMP) pour toutes les femmes était un engagement du Président de la République, un engagement qui trouve dans ce projet de loi des conditions d'application sereines, dignes et sécurisées pour les enfants issus de ce dispositif. C'est tout le sens du travail colossal qui a été mené sur le droit d'accès aux origines et sur l'instauration d'un nouveau mode de filiation. Ce texte permet également d'autres avancées. Je pense en particulier au don d'organes croisé et à l'accès aux transmissions des informations génétiques. Je pense également à l'encadrement des traitements d'intelligence artificielle. Je pense enfin à la gouvernance bioéthique renforcée, qui consolide le débat démocratique. Je sais que certains sur ces travées aimeraient parfois aller plus loin sur certains sujets- d'autres, moins loin -et je respecte ce souhait qui épouse des aspirations sociétales sincères et parfois légitimes. Ce texte ne satisfera pas tout le monde : il sera jugé tantôt frileux, tantôt audacieux. Ce sera toutefois, j'en suis convaincu, un texte équilibré, c'est-à-dire un texte ambitieux sans être aventurier, un texte responsable sans être tiède. Le projet de loi accorde de nouveaux droits et apporte les ajustements rendus nécessaires par les évolutions techniques et sociétales. Accorder de nouveaux droits et de nouvelles protections, c'est la marque d'un progressisme qui a gardé le sens des conquêtes ; croyez bien que je ne perds pas de vue les principes qui donnent toute leur force à ces droits nouveaux. À chaque ligne de chaque article, nous avons scrupuleusement veillé à préserver l'équilibre entre le respect de la dignité de la personne humaine, l'autonomie de chacun et la solidarité de tous. Ces mesures recouvrent notamment, avec l'article 1 du projet de loi, l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules et non mariées. Nous avons pour cela respecté un impératif catégorique : offrir un cadre protecteur pour l'enfant à naître, qui, à sa majorité, aura la possibilité, sans condition, d'accéder aux informations relatives au tiers donneur ainsi qu'à l'identité de ce dernier. Ce cadre protecteur sera garanti par une gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l'Agence de la biomédecine.

ses missions. Nous pouvons être fiers de l'article 1. Je le dis non sans émotion, parce que je pense à tous ces couples de femmes qui, depuis tant d'années, s'engagent dans des parcours du combattant pour mener à bien leur projet parental. Je veux dire à tous ces couples de femmes que, dorénavant, leur projet parental, leur projet familial, sera pleinement reconnu et qu'elles seront accompagnées comme il se doit dans leurs démarches. Il m'est arrivé d'entendre de drôles de propos sur de prétendus « désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ». Par cet article, au contraire, la famille française s'agrandit, dans la diversité de ses modèles et dans la richesse de ses configurations. C'est un enjeu d'égalité ; la force de l'égalité républicaine, c'est précisément de reconnaître la diversité des situations, des parcours et des projets de chacun. Dans le quinquennat précédent, le mariage pour tous a participé de ce mouvement vers l'égalité, bien loin du choc anthropologique redouté par certains. Je rends hommage à tous ceux qui, à l'époque, sur ces travées et ailleurs, ont permis à la France d'être fidèle à sa promesse d'égalité et d'émancipation. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vois aucune raison valable à ce que les équilibres trouvés à l'Assemblée nationale se heurtent à des impasses, ici, au Sénat.

le 21 janvier 2020, nous engagions dans cet hémicycle l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. Près de dix-huit mois plus tard, pour notre troisième rendez-vous sur ce texte, nous ressentons une certaine déception. la navette parlementaire a pu suivre son cours sans procédure accélérée, mais elle n'a pas permis d'enclencher un dialogue constructif entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à tout le moins sur les pans les plus visibles ou les plus importants de ce texte. Il nous appartient aujourd'hui d'en tirer les conséquences. C'est la raison pour laquelle la commission spéciale vous proposera de mettre un terme à nos débats en votant une motion tendant à opposer la question préalable. Cette décision ne va jamais de soi, plus encore quand il s'agit d'une loi de bioéthique : nous le savons, ce n'est pas une loi tout à fait comme une autre. Les lois de bioéthique ont vocation à traduire un équilibre entre ce que la science permet et ce que la société est prête à autoriser. Les enjeux sont aujourd'hui majeurs en matière de recherche, tant l'avancée rapide des connaissances ouvre d'opportunités de mieux comprendre la complexité du vivant. Ce texte est attendu par la communauté scientifique sur ce volet essentiel. Il serait sorti plus fort du Parlement s'il s'était appuyé sur un consensus. À notre regret, cela ne sera pas le cas. Au Sénat, nous avons eu à coeur d'accueillir les perspectives ouvertes par la recherche, notamment sur les cellules souches induites pluripotentes, sans céder sur nos principes éthiques fondamentaux. Ce texte trace en ce sens des avancées dont nous avons soutenu le principe. Nous aurions parfois souhaité aller plus loin, pour ne pas faire prendre un retard préjudiciable à la recherche française dans un environnement international hautement concurrentiel. Nous avons également tenu à affirmer des limites claires. En matière de recherche, notre préoccupation principale a été de veiller à ce que la recherche ne franchisse pas les lignes rouges que sont notamment le respect de la barrière des espèces. Sur les embryons chimériques, les questions soulevées par ce type de manipulation ne peuvent être balayées d'un revers de main et laissées à la seule appréciation de l'Agence de la biomédecine. Sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, nous n'avons pas été suffisamment entendus par nos collègues députés comme par les ministres qui se sont succédé au banc Certes, au terme de nos travaux, nous retenons quelques facteurs de satisfaction. Des propositions issues du Sénat permettront demain, avec l'extension ciblée du dépistage néonatal, de prendre en charge des nouveau-nés sans perdre de précieuses semaines ou années de traitement. Pour autant, le dialogue s'est figé sur des divergences profondes entre nos deux assemblées, comme celles qui portent sur le chapitre relatif à l'assistance médicale à la procréation (AMP). Même sur des points précis comme l'établissement de la filiation ou les modalités de l'accès à l'identité des donneurs de les portes sont trop souvent restées fermées aux propositions de notre rapporteur Muriel Jourda, et ce dès la fin de la première lecture. Et pourtant ... Sur un sujet apparemment moins clivant comme celui de la gouvernance en matière de bioéthique, l'Assemblée nationale a préféré, de la même façon, ne pas tenir compte de nos observations. C'est donc avec regrets, vous l'aurez compris, mes chers collègues, mais en responsabilité, que la commission spéciale vous demandera de voter la motion tendant à opposer la question préalable à l'issue de la discussion générale. Si nous n'avons pu parvenir à un consensus sur ce texte, nos travaux auront contribué à enrichir certains de ses volets.

L'exercice de remise à plat périodique de ces lois est nécessaire du fait de la spécificité de la « matière bioéthique » : son rythme gagnerait à être plus rapide, pour tenir compte de l'évolution rapide de la science et de la société. la définition de ce contenu gagnerait à être moins liée à des calculs politiques. Le texte qui sera définitivement adopté par le Parlement n'est pas parfait. Il laissera aux uns et aux autres dans cet hémicycle, pour des raisons différentes, un goût d'inachevé même s'il trace des avancées. La commission spéciale aurait souhaité aller plus loin par exemple pour valoriser l'acte altruiste de don d'organes, en matière de recherche ou encore, comme l'a défendu notre collègue rapporteur Olivier Henno, pour encadrer l'accès à des tests génétiques déjà présents dans notre quotidien. Sur d'autres points, les garde-fous que la commission spéciale a proposés n'ont pas été retenus par les députés : je le regrette en ce qui concerne le don d'organes des majeurs protégés ou encore le délai de conservation des gamètes de mineurs atteints de pathologie altérant leur fertilité, qu'elle avait proposé d'allonger.

Nous avons également élaboré un dispositif qui permettra d'améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. L'Assemblée nationale a conservé l'ouverture du don du sang aux majeurs protégés, voté dans cet hémicycle, persistant toutefois à refuser le don du sang aux mineurs de 17 ans. Sur les dons de corps, enfin, après les récents scandales, nous avons tenu à prévenir toute exonération générale de responsabilité pénale. Ces avancées issues de nos travaux sont importantes pour la science, pour les patients. Je partage cependant les regrets que Corinne Imbert vient d'exprimer au nom de la commission spéciale que n'ait pu être trouvé un consensus plus large avec nos collègues députés, comme avec le Gouvernement, sur des dispositions plus centrales de ce texte. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules a clivé nos débats, dans cet hémicycle comme dans le cadre de notre dialogue avec l'Assemblée nationale. Que l'on soit favorable- comme je le suis -ou au contraire, comme certains d'entre vous, mes chers collègues, opposé à cette réforme, nous avons été nombreux, dès la première lecture, à regretter l'adjonction de ce sujet à une loi de bioéthique. Cela a éclipsé dans le débat public d'autres enjeux majeurs, et c'est regrettable. Cela a également réduit notre capacité à engager un dialogue serein entre les deux assemblées et à trouver plus d'accord sur les sujets de bioéthique. Après l'échec de la commission mixte paritaire à trouver un accord, principalement en raison des divergences insurmontables exprimées sur ce volet du texte à l'issue de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un texte très proche de ses positions antérieures.

Nous ne pouvons qu'en prendre acte. Mes chers collègues, la commission spéciale vous propose d'en tirer les conséquences en opposant, à l'issue de cette discussion générale, la question préalable. Ce n'est pas l'issue que l'on pouvait espérer pour une loi de bioéthique.

la commission mixte paritaire a échoué et vingt-cinq articles restent en discussion pour la troisième lecture au Sénat du projet de loi relatif à la bioéthique. Nous avons constaté de nombreux points de désaccord ; je le regrette.

une prise en charge totale pour tous par la solidarité nationale, le Sénat a limité le remboursement de l'AMP aux couples hétérosexuels infertiles. À titre personnel, je suis favorable à l'accès de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. En matière de remboursement, j'ai proposé une solution de compromis, avec une prise en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé en cas d'absence de critère médical d'infertilité. Le Sénat a rejeté à deux reprises l'article 2 sur l'autoconservation des ovocytes. Actuellement, en dehors des personnes atteintes de maladies graves, l'autoconservation des ovocytes est uniquement possible en contrepartie d'un don d'ovocytes. Cela ne me semble pas juste. Je suis donc favorable à l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes. Le parcours de l'assistance médicale à la procréation est long et éprouvant.

Je rejoins la position du Sénat sur la question de l'accès aux origines des enfants issus d'un don de gamètes. Je suis favorable à la communication systématique des données non identifiantes, mais à la préservation de l'anonymat des donneurs s'ils le souhaitent. le Sénat avait trouvé un bon équilibre à ce sujet et je regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu cette proposition. En matière de filiation des enfants nés de PMA (procréation médicalement j'approuve la position du Sénat, qui proposait un dispositif d'adoption facilité plutôt qu'une reconnaissance anticipée. Je regrette la disposition, qui, au sein de l'article 4 , marquait une opposition très claire à la GPA en s'opposant à la reconnaissance du père d'intention dans la transcription en France de l'acte de naissance d'un enfant né de GPA à l'étranger. Je suis également très réticent face aux évolutions proposées sur les recherches visant à créer un embryon chimérique ou transgénique. Nous ne maîtrisons pas les risques du devenir des cellules souches humaines humaines introduites dans un embryon animal. Je comprends les enjeux que cette recherche représente en matière de greffe d'organes, mais nous appréhendons cette disposition. La commission spéciale du Sénat, dont je salue le travail, a fait le choix de déposer une motion tendant à opposer la question préalable sur ce projet de loi. Les rapporteurs nous ont fait part de la non-prise en compte des préoccupations du Sénat par les députés.

la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes. Je pense encore à l'accès aux origines pour tous les enfants conçus avec tiers donneur, à leur majorité. Si nous souhaitions aller plus loin sur l'AMP ou dans le traitement de l'accès à l'AMP, en assurant une égalité de traitement au regard de l'identité de genre, il est certain que cette rédaction constitue déjà une avancée sociétale majeure et attendue. L'AMP n'est pas une concession faite à l'époque : elle est l'aboutissement d'un long processus, qui nous amène à reconnaître une liberté, parce qu'elle correspond à une nécessité. Il y a une réalité biologique, mais il y a également une vérité humaine à laquelle nous devons répondre. La société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique, issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts : les deux tiers des Françaises et des Français y sont favorables. Il faut maintenant l'acter. Nous sommes également satisfaits que les députés aient répondu favorablement à un certain nombre de dispositions que nous défendions en deuxième lecture,

regrets. L'Assemblée nationale a maintenu l'article 4 , qui interdit la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger. Cette mesure est à contresens des récentes décisions judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l'étranger ne saurait faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation intégral. Pour ce qui est des modes de filiation, nous privilégions la présomption de parenté pour les couples non mariés, pour le conjoint ou la conjointe, lorsqu'un enfant naît d'une AMP, l'idée étant d'étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. C'est pour nous la solution la plus à même de garantir l'égalité entre les couples. Sur les questions de recherche, nous actons de réelles divergences de fond avec l'Assemblée nationale, le Sénat restant attaché au maintien de l'interdiction absolue de la création d'embryons chimériques afin d'écarter tout risque de franchissement de la barrière des espèces. Cette position est partagée par le groupe Écologiste Enfin, nous regrettons que l'Assemblée nationale n'ait pas voulu profiter de ce véhicule législatif pour clarifier les pratiques et réaffirmer que l'interruption médicale de grossesse (IMG), que ce soit pour raison médicale ou en cas de détresse psychosociale, doit s'appliquer uniformément, dans tous les territoires. On constate encore trop souvent, localement, des divergences d'interprétation quant à l'opportunité de prendre en considération l'ensemble des détresses parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d'une IMG.

Dans nos sociétés contemporaines en mutation, la reconnaissance d'un tel droit est salutaire. Sur ces enjeux, notre boussole est et restera l'humain et l'intérêt supérieur de l'enfant. La parole

sommes une nouvelle fois réunis pour discuter d'un texte charnière pour notre société, je tiens à débuter mon propos en remerciant tous les donneurs mis à l'honneur, il y a deux jours, lors de la vingtième Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs : merci à toutes celles et à tous ceux qui, par leur don ou celui de leurs proches, ont sauvé des vies et qui en sauveront d'autres encore à l'avenir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi relatif cet examen sera court, bien trop court à mon goût. Après une deuxième lecture complexe au Sénat, c'est un rejet simple qui nous attend aujourd'hui. Le texte qui sera adopté définitivement prochainement comprend des avancées majeures et la déception à laquelle invitent nos débats ne doit pas effacer la portée de ce texte. en effet une victoire pour tant de familles, ces familles du XXI siècle singulières et belles. L'ouverture de l'AMP aux femmes seules, aux couples de femmes et aux couples non stériles le démontre. Nous nous félicitons du rétablissement des articles 1 et 2 par l'Assemblée nationale. L'article 4 concernant la filiation des enfants nés à la suite d'une AMP pour les couples de femmes est essentiel pour leur reconnaissance en tant que mères- au pluriel -dès la

de loi permettra à encore plus de parents de remplir une telle mission. L'Assemblée nationale a également rétabli certaines modalités qui nous apparaissent bienvenues.

paires de donneurs et receveurs pour améliorer l'accès à la greffe, à l'article 13, qui permet d'encadrer des dispositifs de neuro-modulation, ou encore à l'article 18, visant à encourager les « passerelles soin-recherches par l'utilisation facilitée d'échantillons conservés à d'autres fins. Le texte répond à l'enjeu unique des lois de bioéthique : amener nos politiques publiques vers l'avenir dans le respect des principes éthiques et moraux qui nous sont chers. C'est là toute la richesse de ces textes, empreints d'une telle complexité qu'ils nous imposent de faire preuve de responsabilité et de bienveillance. Je tiens ici à remercier le Gouvernement de ne pas avoir eu recours à la procédure accélérée. Bien que les débats ne soient pas toujours satisfaisants et que le dialogue s'atténue avec le temps, le texte sort enrichi par ces multiples examens. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail constructif réalisé jusqu'à présent au sein de nos deux assemblées. Toutes les avancées que le texte contient sont nécessaires. Elles répondent aux attentes de nombreux citoyens, aux envies de liberté de tous et au choix de solidarité de chacun. Loin d'être accueilli unanimement, le projet de loi relatif

La majorité de l'Assemblée nationale aurait été intransigeante, nous dit-on. Il nous arrive aussi- hélas ! -dans cet hémicycle de nous heurter à une majorité sénatoriale sûre d'elle et dominatrice. C'est osé ! Pour autant, nous ne renonçons jamais à débattre ni à argumenter pour faire évoluer les consciences. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ! La loi de bioéthique revient régulièrement devant le Parlement pour adapter notre législation aux progrès de la science et à l'évolution des mentalités.

Nous avons foi en la richesse de l'échange, et nous restons ouverts aux évolutions possibles de nos avis par l'expression d'argumentations convaincantes. convaincantes. De faux procès se sont tenus sur des querelles sémantiques qu'il conviendrait de dépasser. On a opposé le droit de l'enfant, avec sa noblesse et son caractère sacré, au droit à l'enfant, qui relèverait d'une exigence malvenue. Comme si le droit à l'enfant n'existait pas

Je trouve également que l'on considère avec suspicion le désir d'enfant des couples hétérosexuels ou homosexuels comme des parents isolés. Faudrait-il avoir honte de désirer un enfant à tout prix ?

Comment pouvons-nous ajouter à cette souffrance physique une détresse morale par le refus d'autoriser le recours aux possibilités thérapeutiques actuelles ? Quel sens aurait le progrès scientifique si l'on en interdisait le bénéfice à ceux qui en ont besoin et qui le réclament ? La finalité ultime de la médecine est de soulager les souffrances. Il faut entendre les souffrances de celles et ceux qui réclament un recours à l'AMP, qu'ils soient en couple hétérosexuel, homosexuel ou, parfois, seuls J'ai aussi entendu parler d'enfant naissant sans père. Un enfant sans père, cela n'existe pas ! Il y a toujours un père biologique. Qu'il soit présent ou non, connu ou inconnu, il existe. Cela ne doit faire aucun doute dans nos esprits, comme dans l'esprit de l'enfant d'une mère célibataire ou d'un couple homosexuel.

C'est la concomitance des deux qui trace la ligne rouge. Je prédis qu'un jour nous aurons à en débattre. Car rien ne sera figé dans le marbre. Heureusement que notre génération ne condamne pas l'humanité pour l'éternité par manque d'humilité. Les mentalités évoluent, comme les techniques. Et c'est toute la richesse de cette démarche bioéthique que d'être réinterrogée régulièrement pour s'enrichir de l'évolution des consciences. Pour cela, nous ne devons pas être privés de débat

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici enfin arrivés en nouvelle et dernière lecture du projet de loi bioéthique, près de deux ans après le début de son examen.

Je veux le dire ici, j'éprouve une certaine colère lorsque je repense à l'imbroglio du vote du Sénat en deuxième lecture, où la majorité de droite a supprimé le droit à la procréation médicalement assistée (PMA) pour tous les couples de femmes et les mères célibataires. Après avoir accepté l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, mais limité son remboursement par la sécurité sociale en première lecture, la droite sénatoriale s'est radicalisée et caricaturée en deuxième lecture, en rejetant complètement l'accès à la PMA aux couples homosexuels, mais aussi aux femmes seules par une manoeuvre, disons-le, politicienne ! Ce durcissement de la position de la droite sénatoriale a renvoyé une image de notre Haute Assemblée en complet décalage avec le reste de la société, puisque 67 % de nos concitoyennes et concitoyens soutiennent l'élargissement de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Mais le Gouvernement est, lui aussi, en décalage avec la société en refusant d'établir, dans ce texte, dès la naissance de l'enfant d'un couple de femmes une filiation claire et solide en faveur des deux femmes, des deux parents.

Le maintien de deux régimes juridiques distincts pour le mode d'établissement de la filiation entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes crée une discrimination selon l'orientation sexuelle que je tenais à dénoncer. Je regrette également que la technique d'aide médicale dite ROPA (réception d'ovocytes de la partenaire) ait été refusée par la majorité gouvernementale aux couples lesbiens. Cette méthode de fécondation (FIV) est pourtant une solution pour des couples de femmes qui décident d'avoir un bébé ensemble et veulent toutes deux participer activement à la grossesse. Enfin, il est dommageable de devoir attendre encore pour autoriser les personnes transgenres à accéder à la procréation médicale assistée et à l'autoconservation des gamètes. des gamètes. Pour toutes ces raisons, il nous semble qu'un nouvel échange dans notre Haute Assemblée était indispensable. Même si le groupe CRCE est favorable aux rédactions proposées par le Sénat sur la recherche sur les embryons, sur les cellules souches pluripotentes ou encore sur la modification du génome, qui nous paraissent plus protectrices contre le franchissement de la barrière des espèces, nous voterons contre la motion de la droite déposée au nom de la commission spéciale, car nous savons qu'elle est essentiellement liée à une opposition à la PMA. À deux jours de la « Marche des fiertés », je veux dire aux couples de femmes, souvent déçues et impatientes, que cette fois-ci, ça y est, la loi va enfin être définitivement adoptée : l'Assemblée nationale aura le dernier mot, et, pour une fois, je ne le regrette pas Après tant d'hésitations, de renoncements, la PMA pour toutes sera autorisée en France. Le camp des progressistes a gagné contre celui des rétrogrades, ... Ça suffit ! ... qui craignent que la société ne s'effondre faute de figure paternelle. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour mettre un terme aux discriminations et aux violences dont sont victimes les personnes LGBTI+.

D'ailleurs, je tiens à remercier nos rapporteurs, qui, tout au long de la navette, n'ont pas manqué d'apporter l'éclairage et les précisions nécessaires à la bonne tenue de nos débats.

Cette déception rassemble l'ensemble des sénateurs tant elle reste vraie, y compris pour ceux qui estiment que le volet sociétal de ce texte n'y avait pas sa place.

Beaucoup de choses ont été dites durant la navette. Les articles ont été largement commentés. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur ce qui a déjà été longuement débattu. longuement débattu. Les divergences irréconciliables concernent les articles 8, 9 et 10, relatifs aux conditions de réalisation des examens génétiques et de communication de leurs résultats à l'intéressé et à sa parentèle, mais aussi les articles 14 et 15 ou encore l'article 17, qui n'interdit la création d'embryons chimériques que lorsqu'ils résultent de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces. Toutefois, d'autres articles ont fait l'objet de rapprochements entre les deux chambres. Ainsi, l'Assemblée nationale a conservé partiellement l'un des apports du Sénat à l'article 7 , qui ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance. À l'article 7 , elle a approuvé la position du Sénat relative à l'encadrement du don de corps. L'article 19 , introduit par le Sénat, a été validé par les députés ; il concerne la réalisation en première intention d'un examen génétique chez les nouveau-nés dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies génétiques ciblées susceptibles de mesure de prévention ou de soins. Les députés ont également suivi le Sénat à l'article 19 sur le diagnostic prénatal et à l'article 23 sur la revalorisation du rôle des conseillers en génétique. Malheureusement, ces points d'accord ne pèsent pas lourd. Qui plus est, le projet de loi n'a pas permis de simplifier et de clarifier la gouvernante de la bioéthique.

commission mixte paritaire non conclusive, et à l'instant où nous nous apprêtons à adopter une question préalable, nous nous interrogeons sur notre capacité à faire entendre notre voix. Tel est pourtant le cadre que nous impose la Constitution, et le phénomène est renforcé par le fait majoritaire. Toutefois, l'intelligibilité de nos débats est garantie par leur publication au. À défaut au. À défaut d'avoir pu modifier profondément le dispositif de ce texte comme certains d'entre nous le souhaitaient, il convient désormais, me semble-t-il, de voter en faveur de la question préalable qui nous sera présentée par la commission spéciale

Mais, bien entendu, le fait que le débat ait été si distendu ne nous a pas permis de travailler correctement. Finalement, nous ressentons une véritable déception législative

-et la droite sénatoriale est restée campée sur des positions radicalement opposées. Ainsi que je l'ai indiqué, le choix d'introduire la réforme de la PMA dans le texte viciait totalement toute chance d'aboutir à un consensus. C'est effectivement ce qui s'est passé.

impossible. La majorité du Sénat s'est évidemment engouffrée dans une telle brèche. Personne ne souhaita plus le consensus ; nous l'avons constaté au fil du temps. De fait, l'issue était jouée d'avance,

ouvert et progressiste a vite été rattrapé. En deuxième lecture, nous avons assisté à un imbroglio parlementaire invraisemblable qui s'est traduit par un recul : le vote de l'amendement excluant les femmes seules de la PMA,

Bien entendu, notre groupe aurait souhaité aller plus loin sur l'application du droit commun relatif à la filiation pour les couples de femmes ou sur les possibilités d'autoconservation ou d'utilisation des gamètes. Le sujet a évidemment été occulté. Les questions de bioéthique sont extraordinairement complexes. Elles sont également politiques.

rappelle, la France dispose d'un modèle spécifique en la matière, puisque la législation sur la bioéthique doit faire l'objet de réexamens réguliers. Le projet de loi consacre tout de même plusieurs avancées la levée en matière de don d'organes de certaines contraintes sur le développement du don croisé, l'affirmation d'un statut de donneur d'organes, des clarifications sur l'encadrement de l'IMG ou la création d'une délégation parlementaire à la bioéthique.

sans bouleverser nos valeurs, identifier des risques, instituer des garde-fous, faire avancer les droits de chacun, en particulier ceux des femmes. Pour nous, c'est cela, le rôle du législateur. Tel est notre état d'esprit. Il est très regrettable que le Sénat ne l'ait pas partagé.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de nos rapporteurs, Muriel Jourda, Corinne Imbert, Olivier Henno et Bernard Jomier. Je n'oublie pas le président de la commission spéciale, Alain Milon, qui a animé nos débats. Lors de l'examen des lois de bioéthique, les questions qui se posent à nous touchent à l'intime. En la matière, nul ne détient la vérité. Chacun doit pouvoir exprimer son opinion. La bonne tenue de nos débats au cours des deux précédentes lectures est à souligner. Il est en effet essentiel d'écouter et de respecter chaque opinion, même si j'ai entendu des propos un peu excessifs ce matin. C'est l'honneur de notre assemblée d'avoir permis un débat ouvert sur un sujet aussi complexe. Au sein du groupe Les Républicains, la liberté sur ce sujet est restée totale tout au long des débats. Chacun a pu se prononcer selon ses convictions, ses croyances, son histoire et ses doutes. La nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, conséquence de l'échec de la commission mixte paritaire, nous laisse un goût amer.

il y aura bientôt la GPA. Le principe posé par l'article 1 au nom d'une égalité en matière de droit à l'enfant et à la procréation devrait intellectuellement inclure la gestation pour autrui. l'examen de l'article 1 en deuxième lecture devant le Sénat, M. le secrétaire d'État Adrien Taquet affirmait : « [L]'ouverture de l'assistance médicale à la procréation sera sans incidence sur l'interdiction de la gestation pour autrui, qui est antinomique des grands principes bioéthiques auxquels nous sommes tous attachés. » Aujourd'hui, sans doute. Mais demain On nous expliquera avec la même assurance qu'il s'agit d'une réforme de justice entre les couples de femmes et d'hommes, ce qui pourra s'entendre. Et on nous vendra alors une GPA dite « éthique Toutes les propositions de la commission spéciale en matière de procréation et de filiation ont été écartées par les députés. Tout en actant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, celle-ci avait maintenu le critère médical, notamment d'infertilité d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels,

Promouvoir une égalité totale entre les couples est illusoire. Un enfant aura toujours deux lignées parentales différentes : c'est ce qui l'inscrit dans le genre humain, universellement mixte. On ne peut pas dire à un enfant qu'il est né de deux pères ou de deux mères, même s'il peut effectivement être élevé dans une famille mono ou homoparentale. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la rédaction de l'article 4, relatif la filiation, retenue par notre assemblée en première et deuxième lectures. Nous avions refusé le principe d'une filiation établie sur le fondement de la volonté pure pour les deux mères. Nous avions considéré l'adoption comme l'unique possibilité d'établir une telle filiation. Le Sénat avait également souhaité un contrôle plus strict de la reconnaissance de la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une GPA. Il avait introduit l'article 4 , qui interdit toute transcription complète à l'état civil dans les cas de GPA. La transcription du lien biologique de filiation est établie, mais l'autre transcription se fait par des moyens autres qu'une transmission automatique, c'est-à-dire par l'adoption.

Certes, le donneur n'est pas le parent. Mais faire don de ses gamètes n'est pas un acte anodin et banal ; c'est transmettre une part de sa propre identité. D'ailleurs, les pays ayant levé l'anonymat ont vu non pas une diminution du nombre de donneurs, mais un changement du profil de ceux-ci. En ce qui concerne le don d'organes, de tissus et de cellules, il est regrettable que les positions du Sénat sur le statut de donneur, ainsi que sur l'abaissement de l'âge du consentement pour le prélèvement de cellules hématopoïétiques et sur les dispositions relatives aux majeurs protégés n'aient pas été retenues par les députés.

Le Sénat avait trouvé le juste équilibre et évité le risque eugénique, mais l'Assemblée nationale a persisté dans sa volonté d'autoriser la création d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal. À défaut d'encadrement crédible, le Sénat s'était positionné contre cette possibilité lors des deux premières lectures, de même qu'il s'était opposé à la modification du génome d'un embryon humain. Signe de leur obstination à vouloir maintenir des dispositions sans valeur ajoutée, les députés ont réintroduit les six membres supplémentaires issus du secteur associatif au sein du CCNE. Nous allons nous prononcer dans quelques instants sur la motion déposée par la commission spéciale. Le rétablissement par l'Assemblée nationale de la quasi-totalité de son texte, y compris sur des points pourtant non clivants, de plus sa détermination à ne pas tenir compte des propositions du Sénat. Pour toutes ces raisons, une large majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de la question préalable. La discussion

Or force est de constater que cette discussion a assez vite pris fin. J'y vois deux causes majeures

et des dispositions « sociétales », selon l'expression consacrée. Évidemment, nous pensons tous aux dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation et en particulier à son extension aux couples de femmes et aux femmes seules.

bouleverser la société, ou à faire état de l'opinion d'une majorité parlementaire. Elles ont vocation à constater un état de la société et à le traduire dans la législation.

Je dis bien « nous devions », car la majorité sénatoriale défend une motion tendant à opposer la question préalable. Celle-ci sera vraisemblablement adoptée, ce qui entraînera le rejet du texte. Je regrette ce choix. Je le regrette, parce que ce texte porte en lui des avancées nécessaires et importantes. Je le regrette surtout, car au-delà des désaccords qui nous opposent le Sénat se prive de débattre sur un texte important, qui intéresse les Français au regard des nombreux sujets de société qu'il traite.

se sont déroulés au premier semestre de 2018 : les citoyens, les associations, les courants de pensée philosophiques ou religieux, les professionnels de santé et les experts scientifiques ont participé aux réflexions. Dans chaque territoire, des débats ont été organisés par des espaces de réflexion éthique régionaux autour de neuf thématiques identifiées par le CCNE. Nous les retrouvons, en grande partie, dans ce texte. Ce projet de loi, je le répète, traite de sujets de société majeurs. Je pense à l'accès aux origines de l'enfant né d'une aide médicale à la procréation avec tiers donneur, ainsi qu'à la gestion des traitements de données relatifs aux tiers donneurs, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons. Je pense également à des sujets complexes, comme l'autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je pense bien sûr à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et à sa prise en charge par l'assurance maladie, avancée sociétale majeure qui figurait dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Sur ce dernier point, pourtant central, comment expliquer les volte-face de la majorité sénatoriale entre la première lecture, où elle avait adopté les dispositions relatives à la PMA, même si elle avait limité son remboursement par la sécurité sociale aux seuls cas d'infertilité,

Vous appelez l'exécutif à la raison ! Pour ma part, je vous invite au respect du débat démocratique et de notre prérogative d'examiner, de construire et de voter la loi

de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, sans même parler de la suppression de l'article 1 de la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité, qui vidait de sa substance ce texte tant attendu par les Français. motions, les unes après les autres, limitent nos débats et notre rôle démocratique. Celle que vous présentez aujourd'hui se justifie, selon vous, par le fait que « le dialogue entre nos deux assemblées n'a jamais eu lieu ». Je n'énumérerai pas de nouveau les apports que vous avez mentionnés dans l'exposé des motifs de cette motion. Mais je me dois d'en citer quelques autres la possibilité d'actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l'accueil d'un embryon dans les établissements chargés de mettre en oeuvre cette procédure le principe selon lequel un employeur ne peut pas proposer la prise en charge des frais d'autoconservation ; la possibilité de préciser les conditions de conservation des gamètes en cas de décès

Il ne s'agit évidemment pas d'être d'accord sur tout, mes chers collègues. Les désaccords sont légitimes, c'est le propre de notre démocratie, sur ces sujets sociétaux et de bioéthique, éminemment complexes, qui touchent à nos consciences individuelles et engagent notre conception même de la société française et de son évolution. Ces divergences d'opinions traversent les groupes politiques, au-delà des clivages traditionnels. Ils touchent à l'intime et parfois même à notre histoire personnelle. Mais le débat renforce les décisions collectives ; c'est par la confrontation des visions que nos sociétés évoluent. Ces points de vue divers sont présents au sein même de notre groupe ; nous les accueillons avec bienveillance. Nous laissons donc chacun libre de son vote et de son positionnement, mais nous restons unis derrière la recherche du dialogue. Alors, faisons honneur à la Haute Assemblée ! Montrons aux Français l'importance du bicamérisme dans notre démocratie ! Soyons à la hauteur des enjeux ! Les questions abordées dans ce projet de loi, quelles que soient nos divergences, sont au coeur de la société et méritent d'être débattues.

masquer cet échec par le vote de cette motion de procédure, mes chers collègues ; vous en assumerez la responsabilité. Pour notre part, nous avons été constants sur ce texte : oui au droit des femmes, oui au progrès de la recherche scientifique, non à cette confusion

tant les divergences sont grandes entre l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale. Il était assez évident que nous n'aboutirions pas. En revanche, nous

d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.